Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la réindustrialisation demeure un objectif essentiel pour la création d’emplois et le recouvrement de notre souveraineté nationale.

Sur le fond – je l’avais d’ailleurs personnellement proposé à la commission des affaires économiques il y a quelques années –, je me réjouis que le Sénat s’engage de la sorte dans des contrôles sur le terrain de l’efficacité de nos politiques publiques. Le programme Territoires d’industrie couvre aujourd’hui environ la moitié des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Sa logique de carte blanche aux territoires, fondée sur un pilotage local assuré par un binôme élu industriel, est pertinente.

Nous ne vous en ferons pas grief, monsieur le ministre, et je salue les travaux menés par M. Gueusquin, que j’ai pu apprécier dans le Gers. Ce que nous pouvons en revanche regretter, c’est que vous ayez reconduit le programme en 2023 sans qu’il ait fait l’objet d’une évaluation sérieuse. La Cour des comptes a d’ailleurs publié, à l’automne dernier, un avis sévère sur la conduite du programme, estimant que le bilan publié par le Gouvernement, qui évoquait triomphalement plusieurs dizaines de milliers d’emplois créés, relevait « uniquement de la communication ». Si cette évaluation avait été faite, on aurait constaté que les effets macroéconomiques ne sont pas partout au rendez vous. Les territoires labellisés devaient notamment bénéficier d’un accès privilégié aux outils de droit commun déployés par les opérateurs partenaires, par exemple les accélérateurs de Bpifrance. Or cette priorisation n’a pas eu lieu. avons mené à bien une première évaluation qualitative et territorialisée du programme, avec les outils et les moyens dont nous disposions. Mais il est désormais absolument nécessaire d’intégrer les périmètres des territoires d’industrie dans des outils de suivi plus robustes,

Non seulement l’accès prioritaire desdits territoires aux programmes de droit commun doit devenir effectif, mais il faut aller plus loin : les opérateurs de l’État doivent élaborer un panier de services spécifiquement conçu pour répondre aux problématiques concrètes identifiées à l’échelle locale dans les territoires d’industrie. En effet, nous avons constaté, lors de nos déplacements, que les priorités du programme telles qu’identifiées au niveau national, en matière d’attractivité notamment, ne recouvrent pas complètement les problématiques évoquées sur le terrain : si l’accès au foncier industriel est crucial, il ne fait pas tout. Créer des logements adaptés aux contraintes des alternants et des jeunes actifs, développer des offres de mobilité, monter des programmes de formation loin des métropoles, tout cela nécessite souvent des solutions sur mesure, qui n’existent pas aujourd’hui.

dans le cadre du programme Territoires d’industrie, en revanche, la collaboration est beaucoup plus ténue : ni le ministère de l’éducation nationale, ni celui de l’enseignement supérieur, ni celui du travail ne sont officiellement parties prenantes au programme. Cela se ressent au niveau local, où les actions en faveur de la formation ou de l’accès à l’emploi mobilisent assez peu les rectorats, les universités, les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) ou encore les bureaux de France Travail. Il nous semble donc indispensable qu’un dialogue structuré entre les ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et du travail soit formalisé au niveau national, afin que ces derniers, à leur tour, mobilisent leurs troupes dans les territoires. Enfin, je reviendrai un instant sur le foncier : à Chalon sur Saône, nous avons constaté le succès du réaménagement de l’ancienne friche Kodak, sur 12 000 mètres carrés ; mais ces très grands sites « clés en main » ne sont pas adaptés aux petites entreprises.

autant de ressorts nécessaires pour relever les défis des environnements économiques changeants d’aujourd’hui. Le programme Territoires d’industrie nous apparaît désormais mûr pour franchir une nouvelle étape vers une dimension plus articulée avec la stratégie nationale de politique industrielle, ce qui servirait mieux l’objectif stratégique de réindustrialisation. Nous pensons donc que ce programme doit être pérennisé. Il est peu coûteux pour les finances publiques – quelques millions d’euros seulement. Il ne remet donc pas en cause l’objectif actuel d’économie. Nous recommandons d’y intégrer, à enveloppe constante, le financement de campagnes de détection de projets industriels, celles ci ayant démontré leur efficacité en matière d’impulsion de nouveaux projets. Nous soulignons l’intérêt d’impliquer l’ensemble des acteurs déterminants des territoires, notamment les régions, cheffes de file du développement économique, dont certaines regardent le programme avec circonspection, ou encore les chambres de commerce et d’industrie qui, par leur connaissance du tissu économique local, surtout dans les territoires ruraux, sont en mesure de booster le dispositif en accompagnant les industriels dans la recherche d’aides publiques, tant au niveau local qu’à l’échelle européenne. Nous sommes convaincus que les chambres de commerce et d’industrie ont vocation à être acteurs de ce dispositif. Sur le modèle des « districts » italiens, qui ont inspiré le programme, nous préconisons d’accompagner la structuration de filières locales, car c’est selon nous de la solidité et de l’efficacité du territoire d’industrie. Observant le modèle italien, nous mesurons combien il permet l’organisation de filières territoriales, qui sont devenues un puissant levier de compétitivité permettant de gagner des parts de marché à l’export. Avec un PIB inférieur d’un tiers à celui de la France, l’Italie exporte aujourd’hui plus de biens que la France ! Le territoire d’industrie idéal, c’est donc celui qui réussit à mettre en valeur des stratégies de filières territoriales portées par des acteurs locaux soutenus régionalement, tant publics que privés, et venant conforter une ambition de réindustrialisation

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mesdames, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, l’ambition du Gouvernement, portée par le Premier ministre, le ministre de l’économie Éric Lombard et moi même, est d’accélérer la réindustrialisation de la France. Je considère le ministère dont j’ai l’honneur d’assumer la charge comme un ministère de combat. Ce combat, c’est celui de la reconquête industrielle de nos territoires : un combat pour plus de prospérité, plus de souveraineté, mais aussi plus de cohésion dans nos territoires ; un combat pour faire de nos territoires, en Hexagone comme en outre mer,

Le rapport préconise premièrement de pérenniser le programme au travers de plusieurs actions. D’abord, il serait recentré sur les « territoires porteurs de véritables projets industriels Sur ce point, je rappelle que la sélection des 183 territoires d’industrie s’est faite sur la base de critères objectifs et exigeants. Tous les territoires labellisés sont porteurs d’initiatives et de potentiel. L’expérience montre qu’il n’y a pas de fatalité industrielle pour nos territoires. Sur 183 territoires d’industrie, 150 étaient en déclin industriel entre 2007 et 2020, mais 110 de ces 150 territoires ont réussi à recréer des emplois depuis 2020. Ces résultats montrent que la réindustrialisation est possible dans tous les territoires. Vous proposez ensuite de renforcer le volet « attractivité » du programme. nécessite, il est vrai, un écosystème complet, avec des infrastructures adaptées, des compétences disponibles et du foncier, sans oublier une offre suffisante d’hébergement. Vous soulignez particulièrement l’enjeu de la formation et du développement des compétences, un thème qui m’est cher et qui est crucial pour l’industrie, 70 000 postes y étant encore vacants. L’industrie a le potentiel d’attirer tous les talents et de les valoriser ; je pense bien sûr aux jeunes, mais aussi aux femmes, qui ne représentent aujourd’hui que 28 % des salariés du secteur. Sur ce chantier des compétences, je souhaite, avec mes collègues du Gouvernement, réaliser le dernier kilomètre des réformes de la formation professionnelle et de l’apprentissage mises en œuvre ces dernières années. Certains territoires d’industrie sont particulièrement actifs et innovants en matière de formation et de compétences ; je pense au territoire Lacq Pau Tarbes, qui est aujourd’hui l’un des fers de lance de la réindustrialisation dans l’aéronautique et dans les technologies vertes.

Je sais que cette question est particulièrement chère à un grand nombre d’entre vous ; je rencontrerai prochainement les sénateurs Jean Baptiste Blanc et Guislain Cambier pour échanger sur ce sujet. J’en viens à présent au deuxième axe des recommandations du rapport, qui concerne la gouvernance et le financement. Vous le savez, le programme Territoires d’industrie repose sur un modèle souple et partenarial. Il associe à l’échelon local l’ensemble des parties prenantes, publiques et privées, autour de binômes composés d’un élu et d’un industriel. Les acteurs du territoire s’organisent autour d’un projet et c’est ce projet qui compte, non les structures.

nous allons nous battre. Je sais pouvoir compter sur votre soutien, lors du prochain débat budgétaire, pour consolider ce programme. J’insiste sur le fait que les financements mobilisés sont ciblés et qu’ils donnent des résultats.

programme Territoires d’industrie est un dispositif original, efficace et à présent éprouvé. Sa première phase a permis de confirmer l’intérêt d’une démarche partenariale, associant les acteurs locaux autour d’un projet industriel de territoire. Les retours du terrain ont permis un certain nombre d’adaptations et votre rapport, mesdames, messieurs les sénateurs,

Le Gouvernement dispose pour répondre d’une durée équivalente. Il aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de répondre à la réplique pendant une minute supplémentaire. L’auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute.

priorisation des territoires présentant déjà un terreau favorable et de ceux ayant mis en œuvre une stratégie partagée ; évaluation globale et mise en place d’indicateurs. La réindustrialisation de notre pays est une absolue nécessité pour réarmer notre économie, renforcer notre souveraineté et redynamiser l’emploi dans nos territoires. C’est parce qu’ils ont su conserver une industrie vivace dans leurs territoires que l’Allemagne, l’Italie ou la Suisse ont des taux d’emploi industriel plus élevés que le nôtre. J’appelle votre attention sur deux points particulièrement intéressants pour notre politique industrielle et pour le développement de l’emploi dans nos territoires : le logement et le transport des salariés. Notre pays se singularise en effet par un manque de mobilité professionnelle. Lorsqu’un bassin d’emploi se tarit au profit d’un autre, les travailleurs, notamment industriels, ont du mal à suivre l’emploi tant ils sont captifs, malgré eux, des logements et des transports. Dans notre pays, déménager a un coût exorbitant, surtout pour ceux qui sont propriétaires de leur logement, soit 57 % des ménages. Les causes, nous les connaissons : manque de construction de logements et très forte fiscalité, pour ce qui est notamment des cessions. Pourtant, les entreprises paient le plus souvent le versement mobilité, qui doit servir au transport de leurs salariés, et participent à l’effort de construction, le fameux 1 % logement, pour pourvoir à leur logement.

entravés, suspendus ou reportés, précisément parce que les conditions de logement des salariés ne sont pas réunies. Je pense que nous avons besoin,

la désindustrialisation de ces dernières années, portée par le mythe d’un pays qui pourrait prospérer sans usine, sans production et sans ouvriers, a fragilisé nos territoires, accru notre dépendance aux importations et obéré notre souveraineté économique. Lancé en 2018, le programme Territoires d’industrie va dans le bon sens en coordonnant l’action de binômes élu industriel, sous le pilotage de l’État et de la région, afin de réindustrialiser au plus près de chaque bassin d’emploi.

en portant une attention particulière à la formation et à l’adaptation des compétences au projet ; ainsi nous donnerons nous les moyens de répondre efficacement aux mutations en cours. En effet, les industriels se heurtent aujourd’hui à des difficultés croissantes pour recruter et cette situation devrait s’aggraver d’ici à 2030. Pourtant, les études révèlent que la disponibilité des compétences est un critère déterminant pour décider des implantations industrielles. C’est pourquoi il faut réinvestir massivement dans une culture scientifique et technique en améliorant le niveau en mathématiques, indispensable à la formation des ingénieurs et des techniciens. Or les résultats des élèves français dans cette discipline sont préoccupants. Il faut aussi améliorer la féminisation des métiers de l’industrie. Il est urgent également de redonner leurs lettres de noblesse aux métiers industriels, souvent mieux rémunérés, en renforçant des initiatives comme la Semaine de l’industrie. Celle ci doit être mieux intégrée dans la scolarité, dans toutes les filières, grâce à une mobilisation accrue des enseignants et à des campagnes nationales plus efficaces. Soulignons enfin le rôle essentiel de l’alternance, mais aussi des écoles de production, que vous avez citées, monsieur le ministre, dans l’écosystème des territoires d’industrie. Toutefois, pour des raisons financières, leur pérennité reste fragile. Or renforcer ces structures est primordial pour préserver notre compétitivité industrielle. Aussi, monsieur le ministre, quelle est votre feuille de route pour faciliter l’émergence d’un capital et de ressources humaines qualifiées, indispensables à la réussite de chaque territoire d’industrie ? La

lancé en 2018, le programme Territoires d’industrie a enfin permis de redonner un souffle à l’industrie dans notre pays, après des décennies de déclin industriel et de fermetures d’usines. Disons les faits tels qu’ils sont : de 1970 à 2010, la désindustrialisation a frappé dans toutes les économies développées, mais elle a été particulièrement sévère Entre 1995 et 2017, la part de l’industrie dans notre économie est passée de 17 % à 11 % du PIB. Mais l’industrie n’est pas qu’une affaire de chiffres. Elle est au cœur de la prospérité de nos territoires, face aux multiples défis liés à l’environnement et à notre souveraineté. Depuis 2017, sous l’impulsion du Président de la République et des gouvernements successifs, une dynamique encourageante se dessine. Ainsi, 130 000 emplois ont été créés dans l’industrie, dont 28 000 pour la

Pas moins de 183 territoires d’industrie ont été labellisés pour la période 2023 2027, ce qui a permis de mettre l’accent sur la notion essentielle de territoire. Implanter une usine, c’est bien plus qu’un acte économique : c’est donner de la vitalité à un territoire, c’est renforcer son attractivité en créant une dynamique. Pourtant, mes chers collègues, tout n’est pas simple. Je pense notamment à la contrainte que représente le zéro artificialisation nette. Bien sûr, personne ne remet en cause la nécessité de préserver nos espaces naturels,… Ah bon ? … mais comment concilier enjeux fonciers, construction de nouvelles usines et réindustrialisation ? Enfin, si ce programme est une réussite, c’est aussi grâce à l’implication dans la gouvernance du binôme local composé d’un élu et d’un industriel. Monsieur le ministre, comment cette collaboration a t elle transformé les relations entre acteurs publics et privés dans les territoires concernés ?

On ne peut pas garantir aux investisseurs industriels que la France pourra accueillir de grands ou de petits projets industriels si l’on ne réfléchit pas à un assouplissement de ces contraintes. C’est la raison pour laquelle, afin de concilier la sobriété foncière et le développement économique,

Le manque de direction claire et les errements persistants en matière de pilotage et de coordination sont révélateurs de l’absence d’une vision globale adaptée aux spécificités de chaque territoire. En réalité, monsieur le ministre, pour faire pousser des carottes, il faut avant tout un terreau fertile. Nos industries ont besoin, pour s’épanouir, d’un ensemble de politiques publiques coordonnées à l’échelon local : recherche, innovation, enseignement supérieur, formation, logement, transport, accompagnement financier, urbanisme, politique foncière. Dès lors, nous ne nous ne pouvons nous satisfaire des discours incantatoires de vos prédécesseurs : nous avons besoin de preuves. Qu’envisagez vous concrètement pour remédier aux dysfonctionnements observés par la Cour des comptes ? Comment, dans cette situation politique instable, comptez vous donner à nos entreprises la capacité de se projeter dans le temps long ?

ministre, le programme Territoires d’industrie, qui est peu coûteux, comme l’a souligné la Cour des comptes, produit incontestablement des effets dans les petites et moyennes villes françaises. La coopération et la mobilisation des acteurs locaux, aux côtés des opérateurs de l’État, contribuent à une dynamique de réindustrialisation de nos territoires. Dans ce type de programme, l’enjeu est de définir le juste niveau d’intervention. Nous sommes convaincus qu’associer les élus locaux et les industriels dans une gouvernance publique privée est une stratégie vertueuse permettant de poser des fondations solides. Des entreprises se réinstallent, des emplois se maintiennent et se créent et des collectivités retrouvent une dynamique économique. Oui, l’ambition et la volonté sont présentes : voilà une première victoire. victoire. Il convient à présent d’aller plus loin, en évaluant le dispositif et en priorisant, les territoires d’industrie ne bénéficiant pas tous d’une mobilisation des acteurs et d’une coordination régionale égales. évaluer pour ne pas saupoudrer et pour capitaliser sur les écosystèmes économiques efficients. Il faut aller plus loin également en simplifiant, car il faut bien reconnaître que la complexité du dispositif nuit à son efficacité.

de véritables moteurs de notre souveraineté économique

Bonduelle : 159 emplois supprimés ; Renault Alpine : 350 emplois menacés ; Fonderie de Bretagne : 500 emplois menacés ; Valéo : 868 emplois menacés ; MA France : 400 emplois supprimés ; Impériales Wheels : 176 emplois supprimés Continental Automotive France : 240 emplois supprimés ; Stellantis : 500 emplois supprimés, 600 menacés ; IBM France : 206 emplois Air Liquide : 479 emplois supprimés, 500 menacés ; ExxonMobil : 677 emplois supprimés ; Thales Aliena Space : 980 emplois supprimés ; Sanofi : 300 emplois supprimés ; Vencorex : 500 emplois menacés General Electric : 484 emplois supprimés ; Dumarey : 500 emplois menacés ; Clestra Metal : 125 emplois menacés ; Mahle Behr : 135 emplois supprimés

pour essayer de résoudre les problèmes. Vous avez cité des exemples d’entreprises en difficulté. Sur tous ces dossiers, nous nous sommes battus. Et nous avons connu des réussites. Nous avons sauvé l’entreprise Niche quelques centaines d’emplois. La semaine dernière, j’étais à Arques, dans le Pas de Calais. Nous avons trouvé un plan de financement qui préserve l’outil industriel pour 4 000 salariés.

au plus près des besoins de notre population et des défis de transition à relever. La planification écologique des transformations de l’économie française ne saurait se limiter à quelques de batteries électriques et à la décarbonation énergétique des process. Gardez le meilleur de Territoires d’industrie et donnez suite aux recommandations du Sénat pour les programmes en cours, monsieur le ministre ! Comment comptez vous stimuler les autres territoires ruraux, qui ne demandent qu’à prendre leur part du développement nécessaire à notre avenir collectif,

ou à la décarbonation. C’est l’ensemble de l’activité économique française, sur l’ensemble des territoires, qui doit être revue

depuis trente ans, le poids de l’industrie dans l’économie française et européenne n’a cessé de chuter. L’industrie est pourtant un moteur indispensable de productivité, de croissance et d’innovation. Elle représente un enjeu majeur pour notre économie, pour la cohésion sociale et territoriale de la France, mais aussi pour notre autonomie stratégique et notre souveraineté technologique. Lancé en 2018, le programme Territoires d’industrie avait pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux enjeux de soutien à l’industrie. Présenté comme une stratégie de reconquête industrielle par et pour les territoires, le programme n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les industriels et les élus locaux.

à savoir le bassin industriel historique, la réunion de lancement s’est tenue dès 2023, et de nombreux projets sont en cours. Pour ce qui est du second, territoire rural peu industrialisé, les projets sont là, les industriels sont inquiets, en raison des retards pris et des difficultés rencontrées, notamment pour recruter. Il faut pérenniser le dispositif et le rendre plus opérationnel. Ne faudrait il pas accompagner différemment les territoires historiquement industriels et les territoires Pour que le système soit efficient malgré des moyens limités, il est indispensable de ne pas se disperser, d’associer et d’accompagner tous les acteurs locaux et industriels et de simplifier. Je souhaite ainsi insister sur le besoin de formation et de promotion des métiers de l’industrie. Quelles actions sont envisagées pour que l’absence de personnel qualifié ne freine pas le déploiement des projets ? La parole

Le Nord est une terre d’industrie, et les élus y ont toujours été attentifs, bien avant le lancement du programme Territoires d’industrie. Ce programme a un mérite : afficher le volontarisme politique, rappeler le caractère stratégique du secteur et les enjeux de souveraineté qui lui sont associés. Je souhaite vous interroger sur les enjeux fonciers de la réindustrialisation et sur le portage politique du dispositif. Le foncier, nous le savons, est un acteur clé de la réindustrialisation, mais il n’apparaît pas comme tel dans le programme. La mise en œuvre complexe du ZAN, le zéro artificialisation nette, tétanise les élus locaux.

Nous devons poursuivre et amplifier le mouvement de recyclage foncier. Le projet de loi de finances pour 2025 devra donc être ambitieux ; je pense notamment au fonds vert. Quelle est votre stratégie foncière pour relever le défi de la réindustrialisation ?

Les régions, pourtant cheffes de file en matière de développement économique, sont snobées dans le dispositif. Là aussi, créons des synergies, au lieu de multiplier les portes d’entrée. Dans le département dont je suis élu, le Nord, nous avons montré qu’ensemble, État, collectivités locales, industriels, partenaires sociaux, nous savons construire des réussites industrielles. Toyota Valenciennes est la plus grande usine automobile de l’Hexagone ; elle vient de fêter sa cinq millionième voiture produite depuis 2001. Faire confiance aux territoires, cela fonctionne

nous avons besoin que nos filières industrielles se mobilisent. J’essaie d’accompagner et de structurer le mouvement dans le cadre du Conseil national de l’industrie. J’ai rencontré les représentants des comités stratégiques de filière pour aborder la question des compétences et des formations. Mon action

C’est toute une vallée qui se trouve dans un état d’inquiétude extrême. Cette inquiétude devrait s’emparer de la France entière, tant les enjeux de souveraineté liés à ces usines sont immenses : enjeu de souveraineté industrielle, enjeu de souveraineté sanitaire, enjeu de défense nationale.

par principe, mais parce qu’elle participe de notre souveraineté, en particulier de notre souveraineté énergétique. Nous continuerons donc à rechercher des solutions

Je vous remercie

de sanctuariser des enveloppes financières dans ces territoires, à l’instar de ce qui a été fait avec l’AMI « Rebond industriel », afin d’accompagner les projets structurants d’investissement productif de nos PME qui ne peuvent pas être soutenus dans le cadre du plan France 2030 Je vous remercie

des dispositifs bien particuliers que sont les missions « Rebond ». Ces missions avaient vocation à soutenir la réindustrialisation de territoires confrontés à des restructurations.

Lancé en 2018, le programme Territoires d’industrie a déjà largement achevé sa phase I. Depuis le mois de novembre 2023, sa phase II est engagée et les sélections sont à ce jour terminées.

Le programme a donc été impuissant à créer une véritable dynamique pour l’emploi industriel dans nos territoires, ce qui était pourtant son objectif initial. Le dispositif Territoires d’industrie n’a pourtant pas manqué d’ambition, pas plus qu’il n’a été sous doté ; il a simplement été mal piloté et mal exécuté, dilué sans distinction dans la masse des aides publiques

Monsieur le ministre, pour la phase II, il y a lieu de corriger le tir en urgence ; à défaut, on risque de devoir de nouveau dépenser – j’ose le dire

Par leur formation technique ciblée, effectuée pour deux tiers en atelier, ces écoles répondent en effet de manière efficace aux besoins des industries locales. Nombre d’entre elles ont bénéficié pour leur création de l’appel à manifestation d’intérêt « Écoles de production », ainsi que de contributions de la part des collectivités locales, y compris, dans certains cas, de la région. Cependant, leur soutenabilité financière est loin d’être évidente : les recettes issues de la taxe d’apprentissage et des ventes des productions des élèves ne suffisent pas à couvrir leurs frais de fonctionnement ; de ce fait, la subvention versée par l’État est rendue L’actuelle convention de financement pluriannuelle signée avec le ministère du travail court jusqu’en 2025. Est il prévu de la renouveler, voire de pérenniser la part « État » du financement des écoles de production ? Il pourrait être opportun également de prévoir à cette occasion un accompagnement financier renforcé des écoles de production pendant leur période d’amorçage, le temps de la montée en charge des effectifs et des commandes. En outre, les écoles de production accueillent le plus souvent des jeunes peu adaptés au système scolaire classique, ou qui en étaient sortis, ainsi que des jeunes « fragiles ». Or, pour ces derniers, qui sont souvent issus de milieux très modestes sont sous statut protégé, le coût du logement, et même celui des produits de première nécessité, peut être un obstacle à la poursuite de la formation. Comment mieux les accompagner sur ce point, pour permettre aux écoles de production de jouer à plein leur rôle de cohésion sociale ? Est il envisageable, par exemple, de donner

à l’élaboration de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a donné une reconnaissance aux écoles de production ; et je crois profondément que cette troisième voie entre les CFA et les lycées professionnels correspond à des

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens en préambule à remercier nos trois rapporteurs de s’être frottés avec succès à l’exercice du « contrôle sénatorial de proximité », ou

Le programme Territoires d’industrie se prêtait par excellence à ce type de contrôle. La vigueur et la richesse de nos échanges, où entre la passion que nous avons pour nos territoires, en montrent

territorial, si souvent sous évalué, dans la constitution des dynamiques économiques. Il faut d’ailleurs saluer l’audace de ceux qui ont porté sur les fonts baptismaux ce programme, qui fait un peu figure d’ovni au sein de la gamme des politiques industrielles déployées par l’État.

Ce que je dis souvent pour le logement à propos des « territoires d’accélération » vaut aussi, me semble t il, pour l’industrie. À partir du retour d’expérience de quelques pionniers, c’est désormais tout le territoire français qui doit devenir un territoire d’industrie.

Si le rapport de notre commission recommande la nomination d’un délégué interministériel à la réindustrialisation, c’est non pas pour créer un nouveau comité Théodule, mais bien pour souligner la nécessité d’activer dans un même élan l’ensemble des leviers de réindustrialisation, qui vont du foncier à la formation en passant par le logement et la recherche. Pour conclure, au moment où nous reprenons – dès demain – l’examen du projet de loi de finances, je me dois de souligner que, dans le panel des outils mobilisables en faveur de la réindustrialisation, les politiques publiques de soutien de l’offre demeurent primordiales pour la compétitivité de nos entreprises. Notre commission soutient naturellement sans réserve les efforts de consolidation budgétaire qui Sur les baisses d’allégements de charges, sur la fiscalité, sur les aides aux entreprises, gardons nous toutefois de la tentation de faire payer à l’industrie un prix disproportionné, au risque de casser pour de bon la fragile dynamique industrielle qui s’était engagée depuis quelques années, mais aussi d’assécher les sources de la croissance future.